n’auraient pu être possibles sans l’engagement exceptionnel des professionnels, des volontaires et des bénévoles qui font la force et assurent la résilience de notre modèle de sécurité civile. En outre, l’année 2024 a été marquée par des inondations sans précédent en France. Ces épisodes climatiques soulignent un impératif : celui, pour la sécurité civile, de disposer de moyens humains et matériels adaptés face à la multiplication des catastrophes naturelles. En ce sens, le PLF pour 2025 prévoit une dotation de 861 millions d’euros en autorisations d’engagement Dans un contexte de contrainte budgétaire, et dans l’attente des conclusions des travaux du Beauvau de la sécurité civile, le Gouvernement propose donc pour le programme 161 un budget qui, pris dans sa globalité, apparaît relativement stable par rapport à l’année précédente. Passée cette observation générale, deux éléments sont à retenir concernant l’analyse des crédits. Premièrement, les crédits d’investissement connaissent une baisse par rapport à 2024. Cette diminution est à nuancer pour deux raisons. D’une part, le niveau d’investissement est extrêmement variable d’une année sur l’autre en fonction des commandes d’aéronefs. Or le renouvellement de la flotte d’avions bombardiers d’eau est reporté à l’horizon 2030.

capacités opérationnelles de la sécurité civile, du moins à court terme. Le PLF pour 2025 prévoit ainsi des crédits élevés pour la location d’aéronefs, pour le financement des pactes capacitaires, ou encore pour le renforcement des colonnes de renfort autant de moyens indispensables à la mise en œuvre d’une solidarité nationale face à la double extension, temporelle et géographique, des risques de catastrophes naturelles. J’en viens aux enjeux thématiques du programme. La question des capacités opérationnelles m’amène d’abord à évoquer la situation de la flotte d’aéronefs de la sécurité civile. Si la saison de feux de forêt a été sous contrôle je tiens à souligner le caractère heureux de cette réussite. En effet, l’extrême mobilisation des agents pour les Jeux, doublée d’un taux de disponibilité anormalement bas des appareils bombardiers d’eau, aurait pu mener à des scénarios plus malheureux, avec un risque de rupture capacitaire. Dans ce contexte, mes chers collègues, j’attire votre attention sur trois points concernant les moyens aériens. Tout d’abord, le renouvellement de la flotte d’hélicoptères se poursuit au rythme prévu, avec la livraison des trois premiers modèles H145 d’ici à la fin de cette année. Ensuite, le budget pour 2025 consacre la pérennisation de crédits dédiés à la location d’aéronefs : 30 millions d’euros sont ainsi prévus pour permettre la location de 10 hélicoptères et de 6 avions.

les deux premiers appareils commandés par la France la Commission européenne ne devraient être livrés qu’en 2030, pour des raisons techniques. Il faudra donc composer avec la flotte existante encore au moins cinq ans, Or cette flotte est vieillissante, ce qui contraint à ménager les appareils et risque de nous forcer à faire évoluer la doctrine française de lutte contre les incendies. Mais les moyens de la sécurité civile ne se résument pas aux aéronefs.

suite des incendies de 2022, pour faire face aux feux de forêt, une enveloppe additionnelle de 150 millions d’euros en AE avait été inscrite dans le PLF pour 2023. La promesse semble aujourd’hui tenue : 37 millions d’euros de CP ont été consommés en 2023 ; 29 millions d’euros devraient l’être en 2024 ; 45 millions d’euros sont prévus pour 2025. Malgré quelques retards, ces pactes sont source de satisfaction. Dans un contexte de contrainte budgétaire, la mutualisation des commandes au niveau national a permis de baisser le prix d’achat des équipements d’environ 30 %. Néanmoins, il est important de souligner que les pactes capacitaires, aujourd’hui essentiellement dédiés à la lutte contre les feux de forêt, constituent un dispositif de financement exceptionnel dont les crédits devraient être consommés dans leur entièreté d’ici à 2027. Or d’autres défis s’imposent à nous. Les conclusions de la récente mission de contrôle relative aux inondations survenues en 2023 et au début de l’année 2024, menée par nos collègues Jean François Rapin et Jean Yves Roux, ont ainsi mis en évidence les limites capacitaires auxquelles ont pu être confrontés nos services de secours. Il paraît donc légitime de réfléchir à la mise en place, à moyen terme, de dispositifs de financement dédiés au renforcement des moyens de prévention et de lutte contre les risques d’inondation. Le sujet des inondations m’amène vers celui de la modernisation des systèmes d’information, de communication et d’alerte de la sécurité civile. De fait, les inondations qui ont touché l’Espagne le mois dernier mettent en lumière l’impératif de disposer d’outils de communication et d’alerte à la population pleinement fonctionnels. Je reste donc attentif à l’évolution des projets de modernisation comme NexSIS et FR Alert, ou encore à la possible mise en place d’un numéro unique d’urgence.

Ce cycle de concertation nationale devrait s’achever au printemps 2025 par la présentation d’un projet de loi portant l’ambition de « poser les bases d’un modèle de sécurité civile renouvelé », trente ans après la loi de départementalisation des services d’incendie.

Alors que, l’année dernière, l’augmentation des crédits avait été largement absorbée par les dépenses de personnel, c’est cette année l’investissement immobilier, grand oublié des deux derniers exercices, qui bénéficie, enfin,

Pourtant, nous sommes encore loin des 400 millions d’euros nécessaires et de l’inscription d’une programmation immobilière dans la durée, seule susceptible d’éviter une dégradation irrémédiable du parc et un glissement vers le locatif, qui coûtera plus cher et privera le gestionnaire de ses marges de manœuvre.

Les obstacles financiers et réglementaires restent trop nombreux et la suspension du paiement des loyers de 5 000 casernes aux collectivités, annoncée en octobre en raison des coûts non budgétés liés à la crise en Nouvelle Calédonie et aux jeux Olympiques et Paralympiques, n’aura pas contribué à renforcer la confiance. Au fond, la trajectoire budgétaire de la gendarmerie ressemble à un mouvement de balancier : soit on finance les augmentations d’effectifs en sacrifiant l’investissement immobilier, soit – comme cette année – on fait porter l’effort sur l’investissement en gelant les augmentations prévues par la Lopmi. Ce n’est pas satisfaisant, mais il n’y a pas de solution miracle.

le titre 2 du projet de budget de la gendarmerie apparaît correctement doté, avec une hausse de 83 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour

Ce serait une bonne chose pour maintenir le nécessaire lien de confiance avec les collectivités, à un moment où celles ci sont confrontées à des contraintes financières sans précédent. Le second sujet de préoccupation sur les effectifs est la baisse marquée du budget de la réserve, là aussi en contradiction avec l’objectif, fixé par la loi de programmation, de 50 000 réservistes en 2027. Avec des crédits en baisse de près de 15 millions d’euros, il apparaît désormais difficile d’atteindre cet objectif, que la Cour des comptes jugeait déjà irréaliste dans son analyse de l’exécution budgétaire 2023, sauf à diminuer le nombre de jours annuels effectués, au risque d’un effet délétère sur la motivation des réservistes. La réserve assume pourtant un rôle de plus en plus important au sein de la gendarmerie, assurant la quasi totalité du spectre des missions. Elle est particulièrement impliquée, par exemple, dans la lutte contre l’immigration illégale et clandestine sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord.

avec une organisation de passeurs qui se professionnalise, n’hésitant pas à user de violence ou à se servir d’enfants comme boucliers contre l’intervention des gendarmes. Je forme le vœu, à la suite de votre déplacement sur le littoral du Pas de Calais, que la position du Royaume Uni évolue, en particulier par le rétablissement d’une voie légale La réserve apparaît donc bien comme une composante indispensable à la gendarmerie, y compris dans les conditions d’emploi les plus dures. En conclusion, un point général sur l’exécution de la Lopmi pour la gendarmerie serait bienvenu, alors que nous approchons de la mi afin d’évaluer si les à coups dus aux contraintes budgétaires dans la trajectoire des effectifs ou dans la gestion immobilière nécessitent d’ajuster la mise en œuvre de la vision stratégique initiale. évaluation, notre commission a préconisé l’adoption des crédits relevant du programme 152 de la mission « Sécurités

chers collègues, avant de nous prononcer sur les crédits prévus pour 2025 au titre de la police et de la gendarmerie nationales, il me semble que plusieurs leçons doivent être tirées de l’exercice 2024. J’en citerai trois.

il est possible de sécuriser efficacement l’espace public dès lors que l’on s’en donne les moyens. Ensuite, les forces ont dû faire face à une succession de crises qui a culminé avec les émeutes en Nouvelle Calédonie. Nous devons prendre conscience de la récurrence de ce type de crises et du fait qu’elles représentent toujours un surcoût. À cet égard, il me semble que nous pourrions réfléchir, monsieur le ministre, à la mise en place d’un système de provisions,

Le fait est connu, mais nous devons le garder à l’esprit alors que nous examinons les crédits de la mission « Sécurités ». Dans le contexte du PLF pour 2025, celle ci fait figure de mission préservée. Au vu des enjeux de sécurité auxquels notre pays fait face, c’était indispensable. Ainsi, les crédits prévus au titre de la police et de la gendarmerie nationales progresseraient de près de 1 milliard d’euros par rapport à l’an passé, soit une hausse de 4,2 %, ce qui n’a rien de négligeable. Assurément, ce budget s’inscrit dans la dynamique que nous avons souhaité impulser en votant la Lopmi, dont les objectifs sont globalement respectés. Ce constat peut toutefois être nuancé à deux titres. Premièrement, les schémas d’emplois nuls qui sont prévus marquent un renoncement par rapport à l’objectif fixé dans la Lopmi, qui prévoyait 856 équivalents temps plein supplémentaires cette année. Cela pourrait créer des difficultés à terme, dans la mesure où les objectifs opérationnels posés en parallèle restent inchangés. Je pense notamment à la création de 238 nouvelles brigades dans la gendarmerie. Deuxièmement, les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la police nationale ne sont pas aux niveaux escomptés. La Lopmi n’a pas permis d’enrayer durablement l’effet de ciseaux observé depuis la fin des années 2010 entre la masse salariale et les moyens matériels des forces. Au delà de 2025, des efforts importants et structurels resteront à mener. Je pense en particulier à l’indispensable remise à niveau du parc immobilier de la gendarmerie.

Devant la commission des lois, monsieur le ministre, vous vous êtes engagé à porter ce combat ; soyez assuré que la commission des lois vous soutiendra. Pour l’heure, le fait que ce budget continue d’augmenter malgré la baisse générale qui est imposée aux dépenses de l’État constitue indéniablement un motif de satisfaction. La commission des lois a donc donné un avis favorable sur l’adoption des crédits de la mission « Sécurités

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des lois a donné un avis favorable sur l’adoption des crédits du programme 161, relatif aux moyens nationaux de la sécurité civile. Dans un contexte budgétaire contraint, ce PLF sanctuarise les montants dédiés aux projets structurants du programme et garantit aux forces de sécurité civile les moyens de mener à bien leurs missions. Cette année encore, malgré des feux de forêt modérés, nous avons pu constater le défi que représente le dérèglement climatique pour les acteurs de la sécurité civile. L’extension de la période des feux, ainsi que l’élargissement des zones à risque sur le territoire métropolitain, va rendre nécessaire des investissements massifs, aux niveaux tant national que départemental. De la même manière, l’intensification du phénomène d’inondations qui a mobilisé, des semaines durant, les militaires et les sapeurs pompiers dans les Hauts de France, puis dans les départements du centre est et du sud, témoigne de la transformation du risque climatique et du besoin d’adapter notre réponse à celui ci. Nous saluons ainsi la hausse notable des montants consacrés aux pactes capacitaires. Ils permettront de soutenir les services d’incendie et de secours, tant pour acquérir des camions citernes que pour se doter de moyens de pompage permettant de réagir face à des épisodes de crues d’une durée et d’une intensité inédites. Si ces crédits sont indispensables pour le soutien à l’investissement des Sdis, ils sont néanmoins

la définition d’un modèle de financement crédible au regard de l’intensification des risques. Par ailleurs, la commission des lois a salué la hausse des crédits consacrés au renouvellement de la flotte d’hélicoptères. Alors que nous nous apprêtons à recevoir

La trajectoire d’acquisition définie par la Lopmi sera donc respectée. Ce constat n’est en revanche pas transposable à la promesse d’acquisition de 16 canadairs avant 2027. La faiblesse des crédits dédiés à cet objectif au sein du budget pour 2025 compromet en effet inévitablement le respect des objectifs annoncés par le Président de la République, avec, au mieux, de premières livraisons à compter de 2028. Le renoncement, au cours de l’année, à la commande de deux canadairs hors programme européen est un autre signal d’alerte concernant le respect de la trajectoire définie. Devant les difficultés liées à la situation monopolistique du constructeur, nous ne pouvons que souhaiter que la France parvienne à trouver des réponses, notamment à l’échelon européen, pour éviter de compromettre sa capacité opérationnelle dans les années à venir. Dans l’attente, le maintien des montants dédiés à la location d’aéronefs permettra de garantir la réactivité de la flotte durant la haute saison des feux.

je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de quinze minutes pour intervenir. La parole est à M. Marc Laménie. Monsieur le président,

et de reconnaissance. Hélas ! 2024 n’a pas été qu’une année de célébrations. Les outre mer, particulièrement la Nouvelle Calédonie, ont été le théâtre de violents affrontements. Nous voulons redire ici que nous condamnons fermement le recours à la violence, qui a entraîné la mort de treize personnes, dont deux gendarmes, et plusieurs centaines de blessés. Nous avons une pensée pour eux et pour leur famille. Ces violences, tout comme les dégradations qui les ont accompagnées, sont inacceptables. Les missions de sécurisation et de maintien de l’ordre ont demandé un effort majeur à nos gendarmes et policiers.

de même légèrement inférieure. En outre, les événements exceptionnels que nous avons cités ont entraîné des dépenses imprévues qu’il faudra bien couvrir. Les contraintes budgétaires nous sommes actuellement confrontées sont très sérieuses, mais elles ne peuvent limiter l’exercice des missions régaliennes de l’État. La Lopmi prévoyait une augmentation des recrutements. Le budget que nous examinons examinons les suspend. Cela ne va pas dans le bon sens. Nous devons respecter la loi de programmation et tenir notre engagement de remettre « du bleu » dans la rue. C’est une demande majeure de nos concitoyens, si ce n’est leur principale L’insécurité progresse dans notre pays et il est de notre devoir d’inverser la tendance. La lutte contre le narcotrafic et, plus largement, contre la criminalité organisée sera probablement l’un des grands chantiers des années à venir. La gangrène des stupéfiants ne touche plus seulement des zones bien circonscrites du territoire. Elle s’est tant étendue ces dernières années que même les villes moyennes et les zones rurales sont touchées par des règlements de comptes. des règlements de comptes. Nous ne pouvons plus laisser faire. Dans la lignée des opérations « place nette » qui ont été menées au début de l’année, il nous faut continuer à lutter de manière implacable contre ce qui ronge nos territoires et notre jeunesse. et la police devront continuer à protéger nos concitoyens contre le risque terroriste, contre la délinquance du quotidien, mais aussi contre les débordements qui, quoique imprévisibles, ne manqueront pas de se produire.

À cela s’ajoute que la France, comme tous ses partenaires européens, fait face à une augmentation des flux migratoires, notamment irréguliers. Surveiller les frontières et éloigner les étrangers qui doivent quitter notre territoire sont deux missions qui requièrent de plus en plus de personnel. Nos forces de l’ordre doivent enfin veiller à assurer la à assurer la sécurité routière. Avec des missions aussi vastes et essentielles, il est évident que les moyens des forces de l’ordre doivent être augmentés.

du ministère de l’intérieur. Nous avons l’obligation de poursuivre les efforts entrepris sans relâche depuis plusieurs années. sur 1 000 euros de dépense publique, seulement 23 euros sont dédiés à la sécurité, contre 575 euros aux dépenses sociales. Notre État social est obèse, impotent et inconséquent ; notre budget régalien est quant à lui à l’os, nos Le parent pauvre des dépenses publiques ne peut plus le demeurer. L’urgence sécuritaire, la vie de milliers de Français, la quiétude et le droit à la sécurité de millions d’autres sont en jeu. la France est devenue, si j’ose dire, l’homme dangereux de l’Europe ! Ainsi, l’indice de paix globale, principal indicateur utilisé pour quantifier la sécurité d’un pays classe la France troisième pays le plus dangereux d’Europe. Le risque de terrorisme est parmi les plus élevés et le taux de criminalité organisée y est désormais plus élevé que chez nos voisins d’Europe occidentale. La douce France jadis chantée par Charles Trenet a laissé place à l’ensauvagement massif et au diktat des narcotrafiquants, souvent sur fond d’enclave islamique. Nous ne pouvons pas lutter contre cette nouvelle barbarie avec les moyens et les outils d’hier. Marianne est défigurée et doit retrouver sa dignité. Cela passe par un budget de courage. Oui, la France ne se combat que d’une seule manière : en donnant des moyens aux héros du quotidien, à ces héros anonymes, ces femmes et ces hommes de courage, de désintéressement et de dévouement que sont nos services de sécurité, nos policiers et nos gendarmes. Et si ce budget est marqué par une hausse incontestable des moyens alloués à la sécurité et par la continuité dans la modernisation des forces de l’ordre,

L’absence de moyens humains supplémentaires pourrait à terme s’avérer préjudiciable pour faire face à des missions de plus en plus complexes et nombreuses.

C’est à saluer. Le Gouvernement peut se féliciter aujourd’hui de la récolte du courage semé hier. Mais nous ne remercierons pas nos forces de l’ordre en gelant les recrutements

Or ces infrastructures souffrent d’un sous investissement chronique qui a engendré, selon la commission des finances du Sénat, une dette grise estimée à 2,2 milliards d’euros sur les dix dernières années.

Il illustre une volonté claire : faire de la sécurité un pilier central de nos politiques publiques. Les moyens financiers qui lui sont alloués traduisent une ambition de moderniser et de renforcer l’efficacité des actions de l’État, un impératif face aux nombreux défis qui subsistent. De grâce, ne baissons pas le rythme, car chaque euro d’argent public en moins pour la sécurité est une parcelle du territoire de la République en plus grignotée par les narcotrafiquants, les criminels et les délinquants, qui menacent notre Nation et avancent à grands pas ! La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec l’examen des crédits alloués à la mission « Sécurités » pour 2025, nous abordons une pierre angulaire des fonctions régaliennes de l’État. Ce budget est marqué par une hausse globale des crédits alloués à la police et à la gendarmerie. Il s’élève à 24,3 milliards d’euros en crédits de paiement, soit une augmentation de 1 milliard d’euros par rapport

cannibalisation des dépenses de personnel au détriment des investissements, en particulier dans l’immobilier et les équipements, freine une modernisation pourtant essentielle. événements récents, qu’il s’agisse des émeutes en Nouvelle Calédonie ou des mobilisations exceptionnelles pour les Jeux, ont souligné l’importance de disposer de forces de sécurité bien équipées et bien formées. L’année 2024 a révélé la nécessité d’une provision budgétaire pour mieux anticiper les surcoûts liés aux crises, à l’instar du modèle de la mission « Défense » pour les opérations extérieures. En matière En matière de sécurité numérique, la hausse de près de 49 % des crédits destinés aux systèmes d’information est un progrès important pour lutter contre les nouvelles menaces, mais une coordination accrue et des ressources humaines adaptées L’état préoccupant du parc immobilier de la gendarmerie, avec une dette grise estimée à 2,2 milliards d’euros, illustre les lacunes d’investissement chroniques dont nous souffrons. La solution passe par des innovations financières, comme le recours aux partenariats public privé, pour engager des rénovations structurelles. À ce titre, je tiens à saluer l’engagement pris par le ministère de l’intérieur de permettre à la gendarmerie d’honorer, dès ce mois ci, les 200 millions d’euros de loyers retard dus aux collectivités. Il y va de la confiance entre l’État et les collectivités, qui ont investi massivement pour le maintien des forces de l’ordre sur leur territoire. Dans un même esprit, il est impératif de garantir à nos forces de l’ordre des conditions de travail dignes, en particulier dans les zones rurales et ultramarines. Fruit d’un compromis nécessaire, ce budget n’en traduit pas moins une volonté sincère, celle de maintenir et de poursuivre les efforts engagés afin de garantir et renforcer la sécurité des Français. Nous sommes cependant conscients que, pour répondre pleinement aux attentes de nos concitoyens et aux défis sécuritaires croissants, trois axes mériteront notre attention. au renforcement des recrutements dans les prochaines années pour atteindre les cibles de la Lopmi, avec un calendrier clair et contraignant. Nous devrons ensuite nous attacher à la révision de nos priorités d’investissement, notamment en matière d’immobilier, pour éviter que la gestion de la dette locative n’alourdisse davantage les budgets futurs.

témoigne d’une réelle volonté de soutien à nos forces de l’ordre et de sécurité, dans un contexte budgétaire très contraint. Aussi le groupe RDPI soutiendra t il l’adoption de ces crédits essentiels, afin de conserver la dynamique positive engagée depuis l’adoption de la Lopmi. La parole

du ministère de l’intérieur visant à assurer la sécurité intérieure, à poursuivre l’effort contre la délinquance, à garantir la protection des populations et les capacités de gestion de crise, et à intensifier la lutte contre les incendies et l’insécurité routière. Ces actions fondamentales pour la société sont au cœur des prérogatives de l’État et nous ne devons pas trembler au moment de leur allouer des moyens ambitieux permettant de répondre aux besoins présents et futurs. La trajectoire globale proposée peut paraître insuffisante pour atteindre ces objectifs. Les crédits proposés par le Gouvernement pour 2025 s’élèvent à 17,3 milliards d’euros en CP, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à Toutefois, cette augmentation doit être analysée à l’aune des coupes budgétaires décidées par le Gouvernement et des dépenses exceptionnelles liées au contexte de la crise en Nouvelle Calédonie.

et Paralympiques que des cérémonies du 80 anniversaire des débarquements de Provence et de Normandie, ainsi que de la Libération de Paris. Grâce aux 35 000 policiers et gendarmes qui ont œuvré lors des JOP, sans oublier les 45 000 bénévoles, la ferveur populaire a pu s’exprimer librement et sans crainte pour soutenir tous les sportifs présents. Cette quiétude a eu néanmoins un coût que notre collègue et rapporteur spécial de la mission « Sécurités », Bruno Belin, a estimé à 814 millions d’euros pour la période 2020 2024 pour la police nationale et à concurrence de 327 millions d’euros sur trois ans pour la gendarmerie. Il faut espérer que ces coûts ainsi que ceux qui sont liés aux opérations de maintien de l’ordre en Nouvelle Calédonie, en Martinique et à Mayotte, lesquels s’élèvent à 155 millions d’euros, seront cantonnés au budget 2024.

Dans le projet annuel de performances de la mission ministérielle « Sécurités », rien n’est dit expressément dans les programmes 176 « Police nationale » et 152 « Gendarmerie nationale sur les mesures à prendre pour éviter une nouvelle situation insurrectionnelle, comme celle dans laquelle a été plongée une partie du territoire français et qui a causé plus de 1 milliard d’euros de dégâts.

elles nécessitant une prise en compte dans le projet de loi de finances : garantir l’adéquation de la formation des forces de l’ordre aux contextes émeutiers avant leur déploiement ; se doter des moyens matériels et des équipements permettant de faire face à des contextes émeutiers longs et protéiformes assurer la sécurisation des bâtiments utilisés par les forces de l’ordre et des armureries pour se prémunir de toute prise d’assaut ; consolider et amplifier l’activité des services de renseignement dans le suivi et la connaissance des « quartiers sensibles » et des phénomènes de violences urbaines faciliter le déploiement de la vidéoprotection au sein des communes rurales ou de petite taille ; assurer un traitement judiciaire des violences urbaines efficace en contexte de crise ou d’émeutes. Même si ces prescriptions n’apparaissent pas explicitement

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

la mettre en œuvre, en assurer le fonctionnement au quotidien et partout sur le territoire de la République. Il s’agit là d’un élément essentiel du pacte républicain, donc de l’égalité républicaine. Pourtant, trop souvent, nombre de nos concitoyens

y remédier. Dans ce domaine, la police municipale ne pourra pas tout faire. Les caméras mises en place par les communes

Il réduit par ailleurs les crédits pour la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Le budget de la police judiciaire serait également réduit de 8 %, alors même que le Gouvernement entend faire de la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé une grande priorité. plus incompréhensible que cette réduction s’ajoute aux baisses déjà consenties les années précédentes et à une dévalorisation du travail des policiers et des gendarmes, condamnés à faire de la politique du chiffre en matière de trafic de stupéfiants, politique épuisante, inefficace et insensée.

investir massivement dans la sécurité civile. À l’exact opposé des besoins, le Gouvernement veut massivement couper les investissements dans le domaine de On mettra en tension les canadairs et on aura un pacte capacitaire inadapté à l’ensemble des défis que la crise climatique nous pose inéluctablement. Certes, les jeux Olympiques sont finis, mais tel n’est pas le cas de la crise climatique.

augmente mal l’appareil répressif en baissant le secours aux personnes, alors qu’il faut urgemment une réforme d’ampleur. À l’inverse, la réforme que le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires appelle de ses vœux vise à rétablir la confiance de la population envers les forces de l’ordre. Ce lien

seulement parce qu’elles sont descendues dans la rue pour défendre une cause : tout cela mine le rapport des citoyens avec la police. Parce que la doctrine de maintien de l’ordre que nous utilisons polarise et augmente la violence qu’elle devrait au contraire combattre, il faut remettre la désescalade et le respect de la déontologie au centre. Alors que le maintien de l’ordre est assuré toujours plus par des unités non spécialisées, comme le pointe la Cour des comptes, il faut veiller à ce que les agents qui encadrent une manifestation aient suivi des formations spécifiques. La France a un centre de formation de renommée européenne pour le maintien de l’ordre. Utilisons le davantage. Parce que les unités sont envoyées toujours plus loin pour des opérations, dans des territoires qu’elles ne connaissent pas ou pas assez, nous devons urgemment réinstaurer une police de proximité. Alors que la réponse purement sécuritaire est vaine, qu’il faut des réponses globales pour les outre mer, ce qui permettrait d’éviter des interventions extrêmement coûteuses – 140 millions d’euros –, qu’il faut enfin créer une autorité de contrôle indépendante de la police et de la gendarmerie, capable de sanctionner efficacement la méconnaissance des règles déontologiques, ce budget ne prévoit rien de tel.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain se félicite de l’augmentation des crédits demandés au titre des forces de sécurité intérieure.

Le Gouvernement nous répondra que ce sera compensé les années suivantes, mais le récent rapport de la Cour des comptes sur la situation marseillaise peut nous faire douter de ce qui

Nous avons pris bonne note des annonces gouvernementales faites récemment à Marseille sur le front de la lutte contre le narcotrafic. Pour autant, comment ne pas pointer quelques inquiétudes relevées dans le récent rapport de la Cour des comptes

le vendredi 22 novembre dernier. Voilà qui peut nous éclairer sur l’état de la menace… La Cour des comptes relève à plusieurs reprises les marges de progrès possible en matière de lutte contre le blanchiment, notamment pour les effectifs de la police judiciaire spécialisés dans le blanchiment. Monsieur le ministre, comment comptez vous répondre à cette problématique ? Plus globalement, les investissements, s’ils sont en progression, restent insuffisants, notamment en ce qui concerne le parc immobilier de la gendarmerie, comme l’illustre la situation récemment mise en lumière par la presse concernant des impayés de loyers à des mairies. M. Bourgi l’a évoqué en commission : la Lopmi prévoyait la création de 200 brigades de gendarmerie d’ici à la fin du quinquennat. Sans effort supplémentaire, nous n’y parviendrons pas. Nous présenterons plusieurs amendements consacrés aux zones de gendarmerie. Nous ne pouvons que regretter les coups de rabot portés aux actions mises en œuvre au titre de la sécurité et de l’éducation routières. Du permis à 1 euro par jour aux actions de sécurité routière en outre mer, en passant par les formations des agents de la délégation à la sécurité routière, ce sont autant d’actions d’importance qui seront touchées l’année qui vient.

cette baisse et la mettre en perspective avec l’augmentation substantielle – 140 millions d’euros supplémentaires – accordée à la sécurité civile dans le cadre de la loi de finances pour 2024. C’est à l’aune de cette donnée que le groupe SER a fait le choix de ne pas déposer d’amendements sur ce programme afin de ne pas nuire aux efforts budgétaires consentis en faveur de la police et de la gendarmerie nationales dans le projet

composée de douze canadairs vieillissants, et bien trop souvent défaillants, ce qui a, hélas ! affecté et limité l’action de nos sapeurs pompiers, confrontés à de nombreux feux de forêt à chaque période estivale. période estivale. Si nous avons pu bénéficier du soutien des véhicules aériens de nos partenaires européens ces dernières années, nous ne sommes pas en mesure d’endiguer nous mêmes ces phénomènes, qui devraient se multiplier au cours des décennies à venir, puisque la moitié de nos forêts seront soumises à des risques élevés d’incendies d’ici à 2050.

Afin que nos engagements votés l’an passé soient tenus, il doit désormais être sérieusement envisagé que l’industrie aérienne française produise son propre modèle d’avion bombardier d’eau.

ainsi qu’à une perte de sens de l’engagement et à un épuisement professionnel, notamment en raison de la multiplication des tâches qui leur sont confiées. Le groupe SER souhaite que l’exécutif prenne ce sujet à bras le corps, en permettant la revalorisation immédiate de ces métiers si importants pour le bon fonctionnement de notre sécurité civile. Il forme le vœu qu’une campagne de recrutement soit menée dans les plus brefs délais, afin de garantir une disponibilité accrue de nos sapeurs pompiers sur le terrain, ainsi que le renouvellement des générations dans la profession. Un certain nombre de gratifications et de bonifications pour leur retraite gagneraient également à être mises en œuvre. Enfin, nous devons engager des investissements afin d’adapter nos infrastructures et nos modes de fonctionnement face au changement climatique. Nous le constatons toutes et tous dans nos départements : les inondations et les crues se multiplient et ne sont plus seulement liées aux épisodes cévenols ou méditerranéens dans le sud de la France. Les pluies diluviennes inhérentes à la hausse des températures et la montée des eaux intrinsèque à la fonte des glaces doivent nous inquiéter ; c’est dès maintenant qu’il faut agir. Aussi, si nous ne pouvons empêcher pleinement ces phénomènes d’advenir, nous pouvons cependant en réduire l’impact sur nos populations, en favorisant la formation du personnel de la sécurité civile à ces enjeux, ainsi qu’en injectant davantage de moyens dans la rénovation de nos infrastructures, afin que celles ci soient plus que celles ci soient plus sûres et résistantes face aux intempéries. Nous appelons ainsi de nos vœux la mise en place de pactes capacitaires dédiés à la prise en charge des conséquences de ces aléas climatiques par les Sdis.

Cependant, nous défendrons quelques amendements pour les rendre mieux disants. Nous défendons quelques uns des combats qui sont les nôtres depuis longtemps. Je pense ici à la création d’un nouveau programme pour défendre de meilleures conditions d’accueil des victimes de violences conjugales et sexuelles dans les commissariats et gendarmeries ou encore au renforcement des moyens de l’Office mineurs (Ofmin). Je pense aussi, quelques semaines après la publication du rapport de l’inspection générale de

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au mois de février 2024, le précédent gouvernement a annulé 154 millions d’euros de crédits des budgets de la police et de la gendarmerie nationales. Résultat : au mois de septembre 2024, la gendarmerie nationale a cessé de payer les deux tiers de ses loyers.

je voudrais croire en votre détermination pour venir à bout de la crise majeure qui sévit en Nouvelle Calédonie et à Mayotte et de la crise migratoire, ainsi que pour mener à bien la lutte contre le narcoterrorisme. Pour cela il faudra avant tout gagner les arbitrages budgétaires au sein même de ce gouvernement… ou du prochain. Votre réconciliation avec Philippe de Villiers est un signe, voire une preuve supplémentaire de votre attachement à la France, celle que nous aimons, et aux Français, ainsi que de votre volonté de les protéger. Comment ne pas être déçu et inquiet après votre conférence de presse à Marseille sur le trafic de stupéfiants, au cours de laquelle le mot « expulsion » n’a pas été prononcé ? Vous n’avez même pas évoqué le phénomène de l’immigration, alors que, selon la police marseillaise, 50 % des trafiquants sont des clandestins et 65 % de la délinquance est le fait d’étrangers. C’est faux ! Pourquoi un tel déni ? Les Marseillais attendent de l’ordre dans leur ville. En effet, quand le pire devient leur quotidien, la fatalité s’installe et la soumission et la corruption deviennent des options de vie.

pour la gauche et la racaille d’extrême gauche qui aiment à voir un « problème systémique dans la police » et ne cessent de traîner dans la boue les forces de l’ordre, qui sont en réalité les victimes d’un racisme anti flic, bien réel En définitive, il nous faut mieux payer, mieux équiper, mieux diriger, mieux considérer le travail quotidien de nos forces de l’ordre. Une police promue et protégée, c’est une population et une France apaisées.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2024, le haut niveau d’engagement des gendarmes et des policiers a permis de relever une succession de défis et de crises, à la fois en métropole et dans les outre mer. Nous devons cette réussite à l’extraordinaire mobilisation de nos forces de sécurité intérieure (FSI) et à leur professionnalisme. Le groupe Union Centriste tient à leur exprimer toute sa reconnaissance. Aujourd’hui, nos débats budgétaires s’inscrivent dans un contexte politique et financier inédit. C’est donc avec un esprit de responsabilité qu’il faut rendre des arbitrages forcément difficiles. Je formulerai trois observations. Tout d’abord, nous constatons que nous nous écartons de la trajectoire fixée par la Lopmi.

Ces renoncements interrogent nécessairement notre capacité à créer les 238 nouvelles brigades de gendarmerie promises par l’État sur nos territoires et à faire de la lutte contre le narcotrafic une priorité.

Du côté de la gendarmerie, l’érosion des effectifs dans les brigades territoriales se fait à bas bruit et exige au moins autant d’attention que la création promise de nouvelles unités. devons pouvoir continuer à nous appuyer sur la réserve opérationnelle. Bref, si nous pouvons comprendre la temporisation concernant la création de nouveaux postes,

Il ne peut pas y avoir de liberté sans ordre républicain ; la servitude naît du désordre. Il ne peut y avoir d’égalité si la loi de la jungle s’applique, car c’est le plus fort qui opprime le plus faible. Enfin, la fraternité ne peut naître que s’il existe une concorde civile.

à l’échelle de la police nationale et de la préfecture de police de Paris. Depuis le 1 janvier 2024, dans le cadre de la réforme de la police nationale, une délégation départementale d’aide aux victimes a été constituée dans chaque département. Toutes ces circonscriptions disposent désormais d’un délégué à l’aide aux victimes.

et la prise en charge de la criminalité organisée au niveau central, puis les unités territoriales de la police nationale au niveau de chaque territoire. Il convient donc d’additionner les deux, c’est très clair et très précis.

des casernes. Cet amendement détaillé vise à répondre aux besoins du Comgend afin de lutter efficacement contre la criminalité et la délinquance à Mayotte. Nos militaires ont besoin de se loger, de travailler dans des conditions dignes, de disposer d’un plateau technique et de renforcer leur état major, en le déplaçant.

dont les bureaux et les cellules. Dès lors, l’équilibre financier s’avère difficile à atteindre pour les petites gendarmeries ; à l’inverse, plus le nombre de logements est élevé, plus il est aisé de financer les locaux de service.

Par cet amendement, nous souhaitons aborder la question centrale de la formation des policiers. Je tiens tout d’abord à alerter le Gouvernement sur l’opacité des crédits alloués dans ce domaine, ce qui soulève un véritable problème démocratique. Jusqu’à l’année dernière, il existait une ligne budgétaire permettant, même imparfaitement, d’identifier les dépenses consacrées à la formation des forces de l’ordre. Ce n’est plus le cas dans ce budget pour 2025. Le travail de suivi et d’évaluation du Parlement s’en trouve ainsi entravé puisqu’il sera très difficile de comparer, d’une année sur l’autre, les moyens effectivement mis en œuvre à cette fin. En procédant par recoupement d’informations, il nous semble néanmoins que les moyens alloués ne sont pas au rendez vous. D’ailleurs, l’objectif, fixé les années précédentes, visant à augmenter le temps de formation continue de 50 a disparu. Il nous paraît donc essentiel de renforcer ces crédits pour permettre le recrutement de personnels de haut niveau. Il s’agit d’une condition indispensable si notre ambition est de disposer d’une police nationale de pointe, singulièrement dans le domaine des enquêtes et de la lutte contre la criminalité organisée.

retiré. Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements identiques ? Favorable

par la conférence des présidents. Nous allons procéder à l’examen des amendements portant sur les objectifs et indicateurs de performance de la mission « Sécurités », figurant

à Mme Corinne Narassiguin. Par cet amendement, nous appelons le Gouvernement à prendre à bras le corps le sujet des contrôles d’identité. Si ces contrôles, réalisés chaque jour par milliers, sont sans aucun doute l’acte de police administrative le plus souvent mis en œuvre